La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (texte de la

discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) pour 2023 est parvenue à établir un texte commun. Lors de ses travaux, René-Paul Savary et moi-même avons veillé à rester fidèles à l'esprit de la majorité sénatoriale. Cette réforme, qui, nous le savons, demandera des efforts aux Français, doit atteindre pleinement son but : ramener notre système de retraite à l'équilibre à l'horizon de 2030, afin de garantir sa soutenabilité financière au bénéfice des générations futures. C'est en ayant cet objectif en tête que, tout en inscrivant ses marqueurs dans le texte, le Sénat a veillé, en première lecture, à rester dans une épure financière proche de l'équilibre. René-Paul Savary vous détaillera certains choix de la commission mixte paritaire, qui se traduiront par des coûts supplémentaires pour le système de retraite par rapport à la version du texte adoptée par le Sénat.

En tout état de cause, mes chers collègues, vous retrouverez dans le texte qui vous est présenté les principales mesures que nous avons examinées et adoptées tout au long de la semaine dernière et même, pour certaines, depuis plusieurs années dans le cadre de Je pense naturellement au décalage progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite de 62 ans à 64 ans, ainsi qu'à l'accélération de la réforme Touraine, sur lesquels repose l'équilibre financier de ce PLFRSS. Je pense aussi à la mise en extinction des principaux régimes spéciaux et à la clause dite du grand-père, aux termes de laquelle les personnes embauchées à compter du 1 septembre 2023 dans les entreprises et institutions concernées seront affiliées au régime général pour le risque vieillesse. Je pense également à l'abandon du projet de transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations, qui a été confirmé par la

Je pense aussi pouvoir dire que ce texte a été profondément enrichi jour après jour, au fil de nos discussions. Ainsi, grâce à votre soutien, nous avons concrétisé des demandes formulées de longue date, par exemple pour les sapeurs-pompiers volontaires, les apprentis, les stagiaires, les étudiants, les sportifs ou encore les enseignants du primaire.

mais je suis convaincu que chaque avancée compte et mérite d'être reconnue en tant que telle. Je pense à la création d'une surcote avant l'âge légal pour les mères ayant atteint la durée d'affiliation requise avant l'âge d'ouverture des droits, ainsi qu'à l'instauration d'un CDI senior, portée avec force et conviction par votre rapporteur René-Paul Savary, dans le respect de l'article L. 1 du code du travail, cher au président du Sénat. Je pense également à la création d'une pension de réversion pour les orphelins, en particulier ceux qui sont en situation de handicap, sur l'initiative de Bruno Retailleau

cette question. Je ne nie évidemment pas les désaccords qui persistent, pas plus que je n'occulte l'expression de l'opposition à la réforme. Je suis sûr, à l'inverse, que personne ne contestera que le débat a eu lieu. lieu avec les partenaires sociaux, après quatre mois de concertation qui ont permis de concrétiser des avancées que personne n'aurait pu imaginer voilà seulement quelques mois. Je pense en particulier à l'emploi des seniors et à la prévention de la pénibilité. Alors que nous pensions les positions des uns et des autres irréconciliables sur ce sujet, nous avons su, je pense, les rapprocher.

L'opposition, moins ici qu'ailleurs peut-être, a choisi un autre fil rouge : celui de l'obstruction méthodique, une obstruction qui sacrifie la mission même d'un parlementaire, qui abîme le débat chaque jour un peu plus, une obstruction, enfin, qui aura été assumée dans une confusion inouïe entre la légitimité du Parlement et l'expression de la rue. De manoeuvres en blocages, d'attaques personnelles en comportements violents, nous avons assisté à une dérive, moins ici qu'ailleurs, certes, ... Pas ici ! ... mais avec la même volonté d'obstruction, que je trouve dangereuse. Je veux le dire avec gravité devant vous : la République ne doit pas céder un pouce de terrain face à ces dérives. Nous les combattrons jour après jour, texte après texte. Beaucoup parmi les opposants à cette réforme ont cité Victor Hugo, tout en foulant parfois au pied son sens aigu du républicanisme, lequel aurait fait honneur à nos débats.

recours lors des trois précédentes réformes des retraites au même vote unique pour surmonter l'obstruction. Lors de la réforme dite Fillon, l'examen en première lecture au Sénat a fait l'objet d'un vote unique en juillet 2003. la réforme dite Woerth, le vote unique a été utilisé en première lecture au Sénat en octobre 2010 sur un quart des amendements. Lors de la réforme dite Touraine, enfin, un vote unique a été utilisé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en novembre 2013.

Alors, oui, pour mettre fin à la négation du parlementarisme et garantir la clarté du débat, le Gouvernement a eu recours à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, et cela au neuvième jour de ralentissement, voire de blocage, des débats.

Nous l'avons fait il y a quelques mois avec l'assurance chômage, nous le faisons avec les retraites. Nous allons le faire, surtout, avec le projet de loi sur le travail et le plein emploi qui vous sera soumis dans quelques semaines. Ce texte portera sur des sujets aussi cruciaux que la mise en place de France Travail,

le travail et l'impôt. Ce vote ne vient pas seulement trancher un débat politique et médiatique de plusieurs mois. Il n'est pas simplement le point final d'une séquence difficile, qui, je suis parfaitement lucide, a angoissé et parfois divisé notre pays. également et surtout la réponse à des questions aussi fondamentales que celles que je pose devant vous ce matin. Voulons-nous, oui ou non, garantir à bientôt 20 millions de retraités qu'ils pourront compter sereinement sur une retraite financée et ainsi préserver leur mode de vie, qu'ils n'ont aucune envie de sacrifier ? Pensons-nous que c'est le travail qui crée la prospérité d'une nation, ou bien que c'est l'impôt qui crée la richesse ? Les valeurs et le projet pour lesquels les Français ont élu leurs représentants au Parlement doivent-ils être défendus par leurs parlementaires, au risque sinon d'une fissure encore plus profonde de la confiance entre le peuple et ses élus ? Mesdames, messieurs les sénateurs, je pourrais m'appesantir sur les réponses que le Gouvernement souhaite apporter à ces questions. On les connaît, vos réponses ! Je pourrais vous redire que l'unique raison pour laquelle nous faisons cette réforme, c'est préserver le patrimoine de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et pouvoir leur dire, sereinement, les yeux dans les yeux : vos pensions ne baisseront pas, vos salaires ne diminueront pas, ... Ils n'augmenteront pas

Je pourrais vous dire enfin que, oui, le respect des engagements pris devant les Français est au coeur du pacte entre le peuple et ses représentants. Mais ce n'est pas à vous, ce n'est pas au Sénat que j'ai besoin de le dire : vous avez toujours respecté vos engagements. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas le Gouvernement qui en décide, ce sont les représentants du peuple par leur vote. Votre vote, c'est la démocratie. Celle-ci est à la fois encadrée et garantie par notre Constitution, sans laquelle rien n'est légitime. Notre Constitution est le coeur même du pacte entre les Français et leurs élus, ce pacte qui existe depuis que la France et les Français votent, ce pacte qui a permis des avancées majeures pour les Français, ce pacte qui a conforté à plusieurs reprises la démocratie lorsqu'elle vacillait et que ses institutions ne parvenaient plus à oeuvrer pour le pays. Voilà ce que je tenais à vous dire en préambule de mon intervention, comme marque de respect du Parlement et du Sénat. Je le disais, mesdames, messieurs les sénateurs, ma conviction, c'est que c'est le travail qui crée la prospérité et que c'est donc par le travail que nous devons financer les évolutions de notre modèle social. L'une des évolutions majeures auxquelles notre pays est soumis, c'est l'évolution de sa démographie. Les faits sont implacables : notre pays vieillit et comptera plus de retraités qu'il n'en a jamais comptés. Notre modèle social devra donc financer plus de retraites que jamais. En 2030, nous aurons à payer chaque mois la pension de 20 millions de retraités, soit un quasi-doublement en une génération. Il y avait 12 millions de pensions de retraite à verser chaque mois au début des années 2000. Aucun pays ne pourrait tenir ce choc sans rien faire ! D'ailleurs, presque tous les pays autour de nous ont réformé ou réforment leur système

combattu, et je remercie la majorité sénatoriale d'avoir contribué à le repousser, non pas par idéologie, je le sais, mais par bon sens. Qui seraient les premières victimes des hausses d'impôts ? Les Français qui travaillent dur, qui se lèvent le matin, qui font vivre leur famille et tourner le pays. Taxer les plus riches ? Taxer les grands groupes ? Cela paraît toujours séduisant, mais l'impôt de trop commence par toucher ceux qui sont en haut et finit par frapper ceux qui sont en bas. Voilà pourquoi, avec la majorité sénatoriale, nous avons repoussé avec détermination toute tentative d'instaurer de nouveaux impôts Voilà pourquoi ce texte se fonde sur des valeurs communes : le travail comme condition de la prospérité et la retraite comme horizon bien mérité, après une vie de travail.

il prend ses racines dans des valeurs communes : le travail, la préservation de notre modèle social et le refus de tout impôt supplémentaire. Ce texte, c'est aussi le vôtre parce que vous l'avez voté et adopté

Je pense aussi au compromis trouvé sur le sujet des carrières longues et à la reprise du dispositif proposé par le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Je précise toutefois que nous avons eu des discussions nourries pour affiner ce dispositif. Enfin, je dirai un mot du dispositif de surcote pour les mères de famille, introduit par la commission des affaires sociales du Sénat et bien sûr intégré à l'accord trouvé hier.

et sous réserve d'un nouveau transfert de taux entre la branche AT-MP et la branche vieillesse, l'équilibre de notre système de retraite en 2030 est garanti par le travail du Parlement et par le compromis qui a été trouvé hier. Voilà, mesdames, Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je tenais à vous dire, alors que vous vous apprêtez à voter une réforme importante pour l'avenir de notre pays et pour le mode de vie des Français, en particulier pour nos retraités. Si je devais résumer ce moment en trois mots, je dirais que nous sommes à un rendez-vous important pour nos institutions, pour notre modèle social et pour notre prospérité. pour nos institutions, car elles garantissent à notre pays de continuer d'avancer. Nos institutions, c'est vous, c'est le Sénat, c'est le Parlement, tout le Parlement, rien que le Parlement. Nos institutions, c'est notre Constitution, toute notre Constitution, rien que notre Constitution.

pour notre prospérité, enfin, car le choix que nous faisons est clair : créer de la richesse par l'activité, non pas par la fiscalité ; aller de l'avant par plus de travail, et non par plus d'impôt. Nous sommes au rendez-vous de nos institutions, de notre modèle social et de notre prospérité, mais s'il est un rendez-vous qui compte plus que tout, un rendez-vous que nous ne devons pas manquer, c'est celui que nous avons avec nos ceux qui travaillent et qui veulent continuer de faire vivre leur famille et de faire tourner leur pays sans outrance et sans blocage, ceux qui travaillent et qui veulent continuer de penser à la retraite comme une période bien méritée de leur vie, au cours de laquelle on récolte enfin, sereinement, le fruit d'une vie de labeur. Ce rendez-vous, celui des promesses que nous avons faites aux Français, celui des engagements que nous avons pris et que nous devons tenir, ce rendez-vous, c'est maintenant ! Aussi, il faut voter ce texte, pour continuer d'aller de l'avant. Nous passons

M. le ministre délégué. Comme je viens de l'indiquer dans mon intervention liminaire, cet amendement vise à modifier l'annexe obligatoire présentant les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre par branche des régimes obligatoires de base pour les années à venir. Il s'agit d'un amendement de coordination, dont l'adoption permettrait de tenir compte, en conformité avec le principe de sincérité des lois financières, des impacts financiers des amendements adoptés au Sénat, ainsi que des modifications effectuées

Nos collègues députés, empêchés en première lecture de débattre du recul de l'âge légal, des carrières longues ou encore des équilibres financiers du texte ont cette fois pu le faire, ce qui a permis aux différentes sensibilités de s'exprimer avant de passer au vote. Cela a été rappelé à de nombreuses reprises, le Sénat, soucieux de la pérennité de notre modèle social et de notre capacité collective à en faire bénéficier les générations futures, porte cette réforme de longue date. Les évolutions démographiques et sociales nous y obligent, car l'émergence de besoins sociaux accrus liés au vieillissement, à la santé ou encore à la nécessité d'investir pour notre jeunesse et l'avenir de notre pays ne nous permet pas de dégager de dégager des marges supplémentaires pour le financement des retraites. Comme je l'indiquais dans la discussion générale, consacrer une part très importante de notre richesse nationale aux retraites relève d'un choix implicite, qu'il nous revient aujourd'hui de clarifier, d'interroger et de discuter. Une part des gains d'espérance de vie qui se poursuivent doit être mobilisée pour le bien commun et la consolidation du financement des retraites. Deux autres éléments supplémentaires plaident en ce sens. D'une part, les sexagénaires d'aujourd'hui n'ont que peu à voir avec leurs aînés des années 1950, qui partaient pourtant à la retraite à 65 ans et pour peu de temps. D'autre part, notre système de retraites s'est enrichi au fil du temps de dispositifs de solidarité qui atténuent les inégalités de carrière et corrigent les effets des règles générales pour les publics qui sont les plus vulnérables pour des raisons de santé, de carrière ou de revenus. C'est pourquoi la présente réforme pèse beaucoup moins que les précédentes sur les publics fragiles. Son examen au Sénat a permis de renforcer cette caractéristique. Nous avons voulu prendre en considération la situation de ceux qui ne peuvent travailler plus longtemps, parce qu'ils ont commencé tôt, parce qu'ils sont en mauvaise santé ou parce que leur fin de carrière manque de perspectives. Au-delà des atténuations des effets de la réforme, le texte comporte des avancées pour les apprentis, les stagiaires, les étudiants ou les élus locaux. Il s'inscrit dans une tendance, jamais démentie, d'élargissement et d'enrichissement de notre système social. Finalement, le texte issu de la CMP propose une réforme qui garantit l'avenir de notre système de retraite sans toutefois faire peser l'effort sur ceux qui ne pourraient le supporter. C'est pourquoi le groupe Les Républicains invite le Sénat à le voter et à prendre ses responsabilités avec courage, comme il l'a fait de manière constante. Nous sommes conscients que ce projet de loi marque une étape et qu'il doit s'accompagner de changements profonds dans la prise en compte des salariés les plus âgés. Dans une économie souffrant d'une pénurie de main-d'oeuvre, il est évident que ceux-ci ont toute leur place. Ce chantier est celui des entreprises et des partenaires sociaux avant d'être celui de la loi. Néanmoins, si des changements législatifs se révélaient nécessaires, nous répondrions présents, comme nous l'avons fait pour la santé au travail, l'assurance chômage et toutes les réformes affectant le fonctionnement du marché du travail.

C'est pourquoi, je le dis d'emblée, notre groupe votera cette réforme des retraites. Notre objectif est non pas de vendre du rêve aux Français, mais bien de fonder la politique sur la réalité.

Face à ce constat, qui peut croire que notre modèle social, en l'état, est pérenne ? Il ne l'est pas. Le Gouvernement se devait d'agir. Le choix était binaire. Augmenter les prélèvements revenait à pénaliser le pouvoir d'achat des Français dans un contexte déjà difficile. Accroître le temps de travail restait donc la seule solution réaliste, alors que l'espérance de vie progresse encore. permettra de sauver notre régime par répartition et de préserver le pouvoir d'achat des Français. Nous saluons ainsi le report de deux ans de l'âge légal. Il s'agit d'une nécessité pour l'équilibre de notre système. Nous regrettons toutefois que l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans notre système par répartition n'ait pas été retenu. Il nous faudra à l'avenir réfléchir à cette question. Si de nombreux Français

de porter un amendement visant à favoriser les carrières longues, idée partagée par de nombreux sénateurs. Nous nous réjouissons donc que le dispositif adopté permette à tous ceux qui ont cotisé au moins cinq trimestres avant 21 ans de partir plus tôt, sans avoir à cotiser plus de 43 annuités. Le coût, de l'ordre de 700 millions d'euros à l'horizon de 2030, est important, mais cette mesure a le mérite de donner plus de lisibilité à la réforme et d'en garantir l'équité. C'est la preuve que le compromis et le consensus sont possibles. Par ailleurs, ce texte contient plusieurs mesures de justice sociale. Les régimes spéciaux avaient été conçus à des périodes où les circonstances l'imposaient, en raison de mauvaises conditions de travail. De nombreux progrès ont été réalisés en la matière, ce qui justifie leur suppression progressive. Le régime général apparaît désormais plus juste pour l'ensemble des Français. Nous saluons donc le maintien de cette mesure par la CMP. Nous saluons également la surcote, allant jusqu'à 5 %, pour les mères de famille ayant réalisé une carrière complète. C'était une nécessité. Cette surcote vient combler un manque et rend hommage à ces femmes qui, tout en travaillant pour subvenir aux besoins de leur famille, participent activement à l'éducation de leurs enfants. Il est d'ailleurs juste d'avoir étendu aux professions libérales la majoration de 10 % de la pension à partir du troisième enfant, tout comme il est juste d'avoir intégré les indemnités journalières de maternité dans le calcul de la pension. Nous nous réjouissons de l'adoption de l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF), qui va bénéficier à près de 40 000 personnes par an. C'est un dispositif que nous soutenons et qui va dans le bon sens, même si certains d'entre nous auraient souhaité aller plus loin. De plus, la prise en compte d'une majoration de trimestres au bénéfice des pompiers volontaires représente une avancée tout à fait justifiée, que nous avions nous-mêmes défendue. Sceptiques quant au CDI senior qui a été proposé, nous sommes rassurés de constater qu'il n'a été maintenu qu'à titre expérimental. Cela permettra d'en juger l'efficacité, avant, éventuellement, de le généraliser. Dans le même registre, l'index seniors peut être un atout. Nous ne doutons pas que cette politique volontariste en faveur de l'emploi des seniors trouvera son aboutissement dans la future loi Travail. Les échanges entre les générations sont une richesse pour les entreprises et doivent être encouragés. Ainsi, avec toutes ces mesures, cette réforme est juste et s'inscrit dans le pacte social français. Elle est un moyen de garantir la pérennité de notre système de retraites, ce qui est indispensable.

Ne soutenant pas la première mesure, et constatant que la seconde n'a pas atteint son but, nous remarquons néanmoins que la droite sénatoriale a consenti à abandonner une partie de ses amendements et remaniements du texte pour éviter un 49.3 à l'Assemblée nationale, après avoir consenti au 44.3 au Sénat. Défendue depuis plusieurs années, cette réforme valait bien quelques sacrifices du rôle du Parlement

au prix, pour beaucoup, d'un prolongement du sas de précarité et de pauvreté, d'une explosion des arrêts maladie de longue durée, du chômage ou du basculement dans les minimas, soit un coût social inédit et une fracture sociale approfondie, ignorée par les partisans de la réforme, qui n'ont rien d'autre à proposer qu'un index non contraignant, l'expérimentation d'un CDI fin de carrière, prétexte à de nouvelles exonérations, exonérations, et un peu de surcote, contre la liberté de partir à la retraite. Un point de PIB, vanté à coups de mensonges sur les 1 200 euros et de marchandages entre les droites et le Gouvernement, pour troquer une mesure d'atténuation contre une autre, avec l'objectif partagé de réaliser l'économie des dépenses sociales qui financera,, les nouvelles baisses d'impôts des plus fortunés. Un point de PIB, en imposant une augmentation contrainte de l'offre de travail et la concurrence entre travailleurs pour faire pression sur les salaires, après avoir dérégulé le marché de l'emploi, permis la dégradation des conditions de travail et voté une restriction des droits au chômage. Un point de PIB, à contre-courant, ignorant les transformations sociétales et sociales en cours, la crise de l'attractivité, les vagues de démissions et le ras-le-bol face à la subordination salariale, au manque d'autonomie et de sens au travail. Un point de PIB, que vous grappillez encore sur le travail, aggravant l'inégalité du partage des richesses, alors que la ponction des dividendes explose et capte, justement, de plus en plus de points de PIB. Un point de PIB, parce que vous ignorez la diversité et l'utilité des services non marchands et le logiciel nouveau pour relever les défis sociaux et climatiques de notre siècle.

Un point de PIB, parce que vous êtes prisonniers d'un logiciel productiviste, incapables d'imaginer une prospérité sans croissance, où serait possible, et même nécessaire, une réduction du temps de travail. Un point de PIB, enfin, en bafouant les corps intermédiaires, acteurs représentatifs de la démocratie sociale moderne, en brutalisant le Parlement, en ignorant le refus radical de cette réforme par le peuple français, en l'imposant comme si ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Vous vous trompez ! Votre refus de la solution de cette impasse, à savoir le recours au référendum, est un nouvel aveu de faiblesse. Retirez votre projet ou soumettez-le au référendum, car vous n'avez pas de mandat du peuple français pour cette réforme. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera contre ce texte,

Certains ont remis en cause la légitimité des outils prévus par notre Constitution ou notre règlement intérieur. Mais l'obstruction d'une minorité n'aura pas empêché la majorité d'entre nous, qui souhaitions améliorer ce texte, de faire ce pour quoi nous sommes élus : voter la loi. ! Je me félicite, mes chers collègues, que nous ayons abouti à ce texte, car c'est le fruit du travail parlementaire- le fruit du travail de toutes les sensibilités de notre chambre. En trouvant un compromis, nous avons répondu à la nécessité d'équilibrer notre système de retraite tout en assurant des droits et progrès nouveaux.

sûr ! Oui, mes chers collègues, nombre de nos concitoyens s'épanouissent dans leur vie active. Ils y trouvent un sens et une place dans notre société. Il n'y a pas de déni dans mes propos : certains métiers sont moins épanouissants que d'autres, plus usants et plus pénibles, et il faut donc adapter notre système à ces publics fragiles. C'est ce que nous avons fait dans ce projet de loi.

par l'extension aux professions libérales de la majoration de 10 % de la pension à partir du troisième enfant, ou encore par la prise en compte des congés maternité.

! Nous avons fixé un minimum de deux trimestres de majoration au titre de l'éducation des enfants au bénéfice de la mère. Cette mesure, portée par la présidente Rossignol, protégera de fait les femmes.

Nous avons aussi adopté plusieurs mesures pour rendre notre système plus juste, par une meilleure prise en compte des carrières hachées, le renforcement des droits à la retraite des aidants, l'attribution de la durée d'assurance au titre de l'éducation en cas de décès de l'enfant, l'intégration des périodes d'emploi des stagiaires et des apprentis dans le calcul des droits à la retraite et la majoration pour les sapeurs-pompiers.

Cette réforme permettra également une prise en compte de l'usure professionnelle, par l'élargissement de l'accès au compte professionnel de prévention et par la création d'un fonds d'investissement dans la prévention Ce texte, mes chers collègues, a été considérablement enrichi par le Sénat, ce qui renforce le rôle de notre chambre dans la fabrique de la loi. Notre système par répartition tout entier est bien bâti sur la solidarité solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités. Nous votons pour une société plus solidaire, prospère et pérenne. Devant une réalité démographique qui est implacable, cela a été rappelé, nous faisons le choix de la responsabilité. Face au déséquilibre de nos finances publiques, nous faisons le choix du travail. Confrontés au risque d'une paupérisation sociale, nous faisons le choix de l'équité. Parce que nous valoriserons toujours le travail par rapport à la taxation excessive, notre groupe votera en faveur de ce texte et des conclusions de la commission mixte

des amendements, parce que nous voulions vous pousser jusque dans vos retranchements. Si nous avons agi de la sorte, c'est parce que nous accompagnons le mouvement social et ces millions de salariés qui ne veulent pas du report de l'âge de la retraite. Quant à

messieurs les ministres, mes chers collègues, sans surprise, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur cette réforme des retraites.

vous a fallu moins de temps en CMP pour « dealer » l'avenir de notre pays qu'il n'en a fallu au Sénat pour déposer un amendement de réécriture de l'article 7, qui a fait tomber 1 300 amendements. Nous n'oublions pas non plus que la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale veulent imposer une réforme à laquelle sont opposés 70 % des Français et 90 % des actifs.

À la crise sociale et environnementale, le Gouvernement et les droites parlementaires ont donc décidé d'ajouter une crise parlementaire et une crise démocratique. Vous imposez une régression sociale en ayant recours aux artifices de la Constitution et du règlement du Sénat. Depuis deux mois, le peuple vous dit non. Ils étaient encore des milliers dans la rue hier, pour la huitième fois, pour dire leur refus de votre projet. Nous avons dénoncé votre réforme injuste, inefficace et impopulaire, mais votre obsession s'est transformée en aveuglement. Le texte issu de la CMP acte une réforme profondément injuste, qui va s'appliquer dès le 1 septembre et contraindre des milliers de concitoyens à retarder leur pot de départ à la retraite de deux ans. Le Gouvernement a donc accepté le contrat de fin de carrière des Républicains. En 2006, un contrat du même type avait été instauré, pour un résultat nul. Le Gouvernement devrait mettre autant d'énergie à lutter contre la fraude patronale aux cotisations sociales et contre l'évasion fiscale. Les sommes recouvrées permettraient de financer notre système de retraite, sans imposer deux années supplémentaires de vie brisée. Contrairement aux affirmations du ministre Gabriel Attal, l'équilibre du système de retraite n'est nullement garanti par cette réforme. Il est assuré par la baisse de la subvention d'équilibre de l'État au régime de retraite et notamment par le gel du point d'indice des fonctionnaires et la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Votre dogme libéral vous fait perdre la raison. Ce sont les politiques d'austérité qui ont entraîné le déséquilibre de notre système de retraite. Je rappelle que le Conseil d'orientation des retraites indique dans son rapport que les mesures d'économies sur la masse salariale publique se traduisent « par une détérioration du solde du système ». Les choix réalisés par la droite sous Nicolas Sarkozy permettent aujourd'hui aux parlementaires Les Républicains d'exiger la généralisation de la capitalisation dans notre système par répartition. Le refus de mettre à contribution les plus riches, le refus de mettre à contribution les dividendes, le refus d'élargir l'assiette de cotisation révèlent les intérêts de ceux que vous protégez. Vous avez même refusé l'augmentation de la cotisation employeur, pourtant proposée par le Haut-Commissariat au Plan pour garantir la pérennité du système de retraite. Vous faites passer les intérêts financiers avant la prise en compte de la pénibilité et des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. La suppression des régimes spéciaux offre une vision éclairante de la manière dont vous concevez la prise en compte de la pénibilité des métiers. En conclusion, nous avons assisté à un marché de dupes entre le Gouvernement et Les Républicains, qui ont renoncé à leurs amendements sur les carrières longues et sur la prise en compte des risques chimiques. Vous portez un projet de classe contre les travailleurs et les travailleuses. La fébrilité du pouvoir monte avec la menace

qui vise à les faire travailler jusque 64 ans, bien au contraire. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste s'opposera jusqu'au bout à cette réforme et soutiendra le mouvement social.

l'occasion de saluer et remercier nos rapporteurs de la qualité de leur travail et de leur connaissance du dossier des retraites. Ils l'ont démontrée tout au long du débat, au cours de la CMP et encore à l'instant en commission.

assure la survie de notre régime par répartition. Surtout, il évite à notre pays de s'endetter pour payer ses retraites. Souvent, nous entendons dans cet hémicycle qu'il y a une bonne bonne et une mauvaise dette. Je partage cette opinion : s'endetter pour investir dans la recherche ou les infrastructures- en un mot, s'endetter pour l'avenir et l'innovation -peut avoir une dimension vertueuse. Toutefois, s'endetter pour le fonctionnement, c'est irresponsable ; c'est compromettre l'avenir.

appelons à l'ouverture d'une conférence sociale après le vote de ce texte. Les sujets sociaux qui sont sur la table sont importants et nombreux. Le travail comme valeur ou contrainte- nous en avons débattu ces derniers

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, aujourd'hui, nous sommes appelés à un vote crucial pour éviter d'infliger de nouveaux sacrifices à nos compatriotes

enfin, pour la gauche, en vue d'expier sa faute d'avoir appelé à voter pour le candidat Macron en 2022 et d'avoir voulu empêcher le vote du texte par une tenue parlementaire d'un aussi mauvais goût que ses tenues vestimentaires. En réalité- dois-je vous le rappeler, mes chers collègues ? -, nous sommes des hommes et des femmes libres. Moi, en tout cas, je le suis ! L'exécutif, lui, est piégé, car Bercy a promis cette réforme des retraites à la Commission européenne pour bénéficier du plan de relance et du « quoi qu'il en coûte ». C'était bien, les vacances ? Il est obligé désormais est non pas sociale, mais économique et idéologique. Il la fera sans nous. En tout cas, il la fera sans moi ! Nous voilà livrés pieds et poings liés à Mme von der Leyen et à l'Union européenne, alors que notre participation nette à son budget est de 10 milliards d'euros par an. En voilà des économies

ce n'est pas la faute des Français si, pour se plier aux exigences de l'ultralibéralisme, les gouvernements ont abandonné depuis trente ans notre tissu agricole et industriel à une concurrence étrangère déloyale, jetant des millions de Français au chômage et nous privant ainsi d'autant de cotisants. Reporter l'âge de départ à la retraite, c'est demander plus d'efforts aux Français pour s'éviter de tailler dans les gisements d'économies tabous. En effet, des économies, il y en a à faire, sur la fraude sociale- de 20 à 30 milliards

Comme les précédents, le gouvernement actuel préfère sacrifier les travailleurs et les mères de famille plutôt que son allégeance européiste en engageant les réformes structurelles nécessaires et urgentes. De grâce, revenons à un État stratège, qui protège le présent et prévoit l'avenir en soutenant l'industrie et le monde paysan, créons des emplois qualifiés pour les plus jeunes et engageons une politique familiale ambitieuse encourageant la natalité française, et exclusivement française. de la République fait le tour du monde pour fuir la colère des Français, le Sénat doit lui envoyer un message clair : quand Emmanuel Macron prend une cuite à Kinshasa, ce n'est pas aux Français d'avoir la gueule de bois C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à refuser le grand déclassement, en faisant un bras d'honneur à cet injuste projet de loi.

ainsi allé jusqu'au vote sur l'ensemble, ce que nos collègues de l'Assemblée nationale n'ont pu faire. Cependant, dans notre hémicycle aussi, la forme l'a trop souvent emporté sur le fond, la politesse en plus. Amendements et sous-amendements déclinés à l'infini et petit livre vert brandi très fréquemment : toute la palette des outils de l'obstruction parlementaire a été utilisée. Le Parlement ne sort pas grandi de cet épisode. La réforme méritait des débats plus approfondis sur bien des aspects. Il a fallu en passer par l'article 44.3 pour pouvoir se pencher sur tous les articles. Soyons lucides : une réforme nous semble nécessaire, car la logique démographique à l'oeuvre depuis plusieurs décennies menace l'équilibre financier de notre régime régime de retraite. C'est une évidence. Le système a un grand défaut : il ne supporte pas une donnée pourtant heureuse, celle de l'allongement de l'espérance de vie. C'est cette équation qu'il nous faut résoudre, tout en tenant compte de certaines situations. Tous les métiers ne se valent pas. Ce que certains peuvent faire jusqu'à 64 ans, d'autres ne le peuvent pas. Il y a l'exposition au risque. Il y a les accidents de la vie. Il y a le manque d'offres d'emploi pour les seniors.

Nos collègues sont parvenus à un accord. C'est assez clair, les travaux de la commission portent la marque du Sénat. Bien entendu, les fondamentaux du texte gouvernemental demeurent, dont le fameux article 7 sur l'âge légal de départ, ainsi que l'index seniors, qui avait été réintroduit par notre assemblée. Nos collègues rapporteurs ont exposé les principaux apports de notre assemblée. Je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour saluer les améliorations concernant les carrières longues, mais aussi pour regretter le recul sur l'usure professionnelle à la suite du retrait du critère d'exposition aux agents chimiques dangereux. Mes chers collègues, la balle sera cette après-midi dans le camp de l'Assemblée nationale. En attendant, je ne cacherai pas les différentes sensibilités qui existent au sein de mon groupe. Chacun a voté jusqu'à présent selon ses convictions : il en sera de même aujourd'hui. Tout au long des débats, nous nous sommes toujours rassemblés sur les nombreux défis de la réforme : la pénibilité, les carrières longues, l'emploi des seniors, la compensation de l'engagement citoyen et bénévole, ou encore la possibilité de rachat de trimestres pour différents profils. Une dizaine de nos amendements ont été adoptés, et certains, qui ont survécu à la CMP, visent à répondre à quelques-unes de nos attentes. Je pense aux jeunes en apprentissage, aux étudiants, aux travailleurs handicapés, aux sapeurs-pompiers volontaires ou encore aux femmes, pour lesquelles des aménagements ont été apportés. et Social Européen, c'est l'idée que la solidarité, une valeur républicaine à laquelle nous sommes fortement attachés, continue de guider le régime par répartition que la France a mis en place en 1945 et auquel nos concitoyens restent très attachés.

je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, dans les territoires d'outre-mer subsistent un grand nombre de disparités, notamment du fait de l'éloignement géographique avec la métropole. métropole. La vie y est chère, le chômage y est deux à trois fois plus élevé et le taux de pauvreté avoisine les 40 % en moyenne. Depuis près de vingt ans, les crises économiques et sanitaires s'y succèdent- chikungunya, « gilets jaunes », covid-19, etc. entraînant des conséquences encore plus frappantes qu'en métropole, à l'image de l'augmentation constante des prix, de la suppression de milliers d'emplois ou encore de la diminution du nombre de nouveaux logements construits. Depuis 2019, les effets de l'actuelle crise sanitaire ont accentué le mal-être social, les inégalités et la précarisation de nombreux concitoyens ultramarins. Parmi les très nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est c'est sans aucun doute le logement, au côté de l'emploi, qui figure en haut du classement. Si le manque de logements est malheureusement une triste réalité qui se ressent chaque jour, un phénomène suscite de plus en plus l'inquiétude des pouvoirs publics et des associations de défense de consommateurs : la non-décence des logements sociaux existants. Bien que toute la France soit concernée, l'outre-mer l'est tout particulièrement. Le texte que je vous propose aujourd'hui a d'abord été déposé à l'Assemblée nationale par l'ancien député de La Réunion qui a été comme moi interpellé par la situation préoccupante de notre île. Une très grande partie de notre population est confrontée à des malfaçons et à des problèmes d'humidité ou de sécurité électrique, avec toutes les conséquences qui vont avec, notamment pour la santé. Tant dans les logements anciens que dans les constructions neuves, beaucoup vivent dans des conditions d'extrême insalubrité ou d'indécence. Aussi, cette proposition de loi vise-t-elle à inciter encore plus fortement les bailleurs à mettre en conformité leurs logements avec les critères de décence fixés par la loi.

Le texte de l'Assemblée nationale avait été cosigné par des députés métropolitains comme ultramarins, notamment par deux vice-présidents du parti Les Républicains. Parce que tous les territoires de la République sont susceptibles d'avoir besoin de ce dispositif, nous avions conservé l'application nationale de la proposition. La commission nous a dit qu'une telle application ferait courir le risque d'effets de bord. Pour répondre aux inquiétudes, nous proposons, comme la commission l'envisageait initialement, une expérimentation ciblée sur le territoire de La Réunion. En effet, si le problème du logement non décent ne se pose pas qu'à La Réunion, il s'y pose là-bas avec beaucoup d'acuité. La commission a alors estimé qu'une telle expérimentation ferait courir le risque d'une rupture d'égalité. Pour nos concitoyens qui subissent le mal-logement, pour tous ceux qui vivent dans les moisissures, dans l'inquiétude d'un dégât des eaux ou d'un accident électrique causé par les infiltrations ou les malfaçons, je ne puis me résoudre à ne rien faire. Tout comme six députés sur sept de La Réunion, tout comme mes trois collègues sénateurs de ce département, j'observe régulièrement la situation de notre territoire. Des personnes âgées, d'autres en situation de handicap, des familles nombreuses déjà durement touchées par la précarité financière, énergétique et sociale vivent dans des conditions parfois dignes du tiers-monde, alors que nous sommes au XXI siècle et dans un pays qui figure parmi les premières puissances mondiales. Nous ne pouvons pas rester sans solution. Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Si la route est encore longue avant de résoudre toutes les difficultés qui sont au coeur du problème du logement dans nos territoires, je veux faire ce premier pas avec vous. Il consiste à empêcher que l'on puisse tirer profit des infractions à la loi. Un bailleur qui met en location un logement non décent ne doit pas toucher de loyers. Il ne s'agit pas d'exempter le locataire du paiement, puisqu'il devra continuer de le verser. Mais le bailleur ne percevra les loyers que lorsqu'il aura mis son bien en conformité avec les critères de décence fixés par la loi. Afin de permettre un suivi de cette loi, je proposerai qu'une commission mixte soit mise en place sur le territoire réunionnais, composée à parité de membres de la société civile et des institutions publiques nommés par décret ministériel, afin

En votant aujourd'hui cette proposition de loi, nous mettrons les choses en mouvement. Nous permettrons à la navette parlementaire d'enrichir le texte. Nous affirmerons aux bailleurs notre détermination à faire respecter la loi. Cette mobilisation, à laquelle je vous appelle aujourd'hui, mes chers collègues, représente un pas supplémentaire pour faire de la lutte contre le mal-logement une priorité politique essentielle, afin de répondre aux besoins des citoyens mal logés, en souhaitant que toutes les collectivités puissent à terme porter cet enjeu crucial à la bonne échelle. Il s'agit simplement de garantir le respect d'un droit fondamental pour permettre à chaque citoyen d'accéder à un logement digne et décent adapté à ses besoins et ses ressources et de s'y maintenir. Cette proposition de loi est une réponse qui devra incontestablement en appeler d'autres. d'autres. Une réflexion beaucoup plus large devra ainsi être menée, particulièrement dans les outre-mer, notamment sur les questions de production de logements sociaux et de lutte contre le sans-abrisme. Je demande à l'État de prendre toutes ses responsabilités et de faire de la lutte contre le mal-logement une grande cause nationale. L'abbé Pierre disait : « La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société est l'indifférence ».

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question du logement non décent est malheureusement un sujet récurrent dans notre hémicycle. Les chiffres montrent que nous n'avons pas encore trouvé les clés pour résorber ce fléau en France, il y aurait au moins 420 000 logements indignes. Outre-mer, la situation est encore pire : il n'y en aurait pas moins de 110 000 dans les départements et C'est dix fois plus qu'en métropole ! À La Réunion, le département de Jean-Louis Lagourgue, il y en aurait 18 000. C'est pourquoi je voudrais doublement remercier Jean-Louis Lagourgue : tout d'abord, pour attirer de nouveau notre attention sur la situation de ces ménages qui sont confrontés à des conditions de vie vraiment dramatiques, ensuite, pour nous permettre de nous focaliser sur la situation particulièrement dégradée du logement en outre-mer. J'en avais déjà dressé le constat il y a un an et demi, dans le rapport d'information sur la politique du logement en outre-mer que j'ai cosigné avec nos collègues Guillaume Gontard et Victorin Lurel au nom de la délégation sénatoriale C'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur, car, au-delà du seul aspect matériel, la dégradation de l'habitat a des répercussions sur tous les aspects de la vie de ses occupants : ce sont des problèmes respiratoires causés par des moisissures, c'est un jeune qui ne peut pas s'isoler pour faire ses devoirs à cause d'une fuite dans le plafond, Face à ces problèmes, les locataires se sentent souvent démunis. Pour lutter contre l'habitat dégradé, le dispositif proposé est simple et, je dois le dire, séduisant prolonger le dispositif actuel de retenue temporaire des allocations de logement, lorsque le logement est déclaré non décent, en consignant le reste à charge du loyer. est de faire pression sur les propriétaires, pour qu'ils engagent rapidement les travaux de mise en décence nécessaires. Je vois cependant plusieurs écueils à la mise en oeuvre de ce dispositif. Tout d'abord, la notion de non-décence ne s'applique, en droit, qu'aux logements locatifs. Le problème des propriétaires occupants de logements insalubres ou indignes ne fait donc pas partie du champ de la proposition de loi. Or ils sont nombreux, particulièrement dans nos outre-mer. Ensuite, le dispositif proposé ne concerne que les locataires qui bénéficient d'allocations de logement. C'est donc une petite partie du logement dégradé qui pourrait, en théorie, être traitée par le dispositif proposé. Or, pour cette petite part, la procédure actuelle de retenue des allocations de logement est déjà très efficace : selon les services de l'État, plus de 95 % des procédures engagées aboutiraient à une remise en état dans les dix mois prévus. Surtout, tous les acteurs que j'ai interrogés m'ont fait part de leurs craintes quant à des effets de bord négatifs, à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. En ce qui concerne les propriétaires, je voudrais d'entrée de jeu souligner que les possesseurs de logements non décents ne sont pas tous des marchands de sommeil, loin de là. Les critères de non-décence ont été considérablement renforcés ces dernières années. C'est bien entendu une très bonne chose, mais le sens juridique du mot « décence » s'est ainsi beaucoup éloigné de son acception courante, ce qui brouille quelque peu les repères.

D'ici à 2034, c'est l'ensemble des logements classés E, F et G qui seront qualifiés de « non décents ». Cela rend nécessaire la rénovation de dizaines de milliers de logements locatifs, ce qui représente des investissements considérables pour les propriétaires. Serait-il raisonnable de les priver, précisément maintenant, d'un complément de revenu qui pourrait justement financer ces travaux de mise aux normes ? Dans une perspective plus large, ce ne serait d'ailleurs pas forcément rendre service aux locataires d'ores et déjà, on constate une surreprésentation des passoires énergétiques dans les mises en vente de logements. Ce sont autant de logements qui sortent du parc locatif, temporairement ou définitivement. Or la tension du marché locatif peut aussi favoriser, indirectement, le maintien dans des logements non décents, lorsque les prix pratiqués sont trop élevés pour que les locataires osent quitter leur logement ou même tenter de faire valoir leurs droits auprès des bailleurs. En outre, introduire une procédure active de consignation du reste à charge pourrait, si cette procédure était mal comprise par les locataires, amener une partie d'entre eux à cesser purement et simplement de payer leur loyer. Ils se mettraient ainsi en tort et s'exposeraient à une expulsion. Aussi, loin de protéger les locataires, le dispositif risquerait de les fragiliser encore davantage. En réalité, la question de la résorption du logement non décent nécessite de prendre en compte tout l'écosystème du logement. Il faut évidemment mieux informer les locataires sur leurs droits. Il faut les encourager à activer la procédure existante de retenue des allocations, qui, je le répète, est très efficace, et les encourager à aller devant le juge pour obtenir une injonction à réaliser des travaux, voire une diminution du loyer si le logement demeure non décent. Il faut également mieux accompagner les propriétaires, notamment en faisant connaître les aides à la rénovation- elles sont nombreuses. Je comprends le sentiment d'urgence qui sous-tend cette proposition de loi, particulièrement dans nos outre-mer. Mais à l'écoute de mes interlocuteurs réunionnais, j'ai surtout compris que le sujet dépassait largement le champ de l'habitat indécent : la plupart des cas évoqués lors des auditions relevaient clairement de l'habitat indigne ou insalubre, voire de situations de péril. Or, pour ces situations, il existe d'autres procédures, bien plus rapides et plus coercitives, pour contraindre le propriétaire à faire des travaux, voire les réaliser d'office. Que ces procédures ne soient pas mises en oeuvre par les autorités administratives, qui en ont le pouvoir en temps utile, c'est un autre problème ... On m'a aussi parlé d'immeubles de moins de dix ans tenus par des étais, de bâtiments soudainement sortis « non décents » d'une opération de réhabilitation ... Ce sont les symptômes de problèmes systémiques du secteur du et du logement à La Réunion : nombre trop limité d'entreprises de taille critique ; difficultés d'approvisionnement en matériaux de qualité ; déficit d'encadrement intermédiaire des chantiers et de contrôle qualité ; rigidité du mécanisme de la garantie décennale Sans parler de l'inadaptation de certaines normes aux territoires ultramarins. En résumé, pour élaborer des stratégies efficaces de lutte contre l'habitat dégradé, que ce soit en métropole ou outre-mer, c'est l'ensemble de l'écosystème qu'il faut prendre en compte, et pas simplement la relation contractuelle entre les locataires et les bailleurs, qui sont en bout de chaîne et pâtissent de ces situations. Pour toutes ces raisons, la commission n'est pas favorable à cette proposition de loi. La parole

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat doit aujourd'hui s'exprimer sur la proposition de loi du sénateur Jean-Louis Lagourgue visant à mieux protéger les locataires bénéficiant d'une allocation de logement et vivant dans un habitat non décent. Dans son article unique, ce texte vise à augmenter la contrainte qui pèse sur les propriétaires bailleurs en vue de procéder aux travaux de mise en décence des logements loués à des personnes bénéficiant des APL. Même si le Gouvernement partage pleinement l'objectif de cette proposition de loi, nous constatons que le mécanisme actuel de conservation des aides est suffisant pour mettre fin aux situations de non-décence. À ce jour, la plupart des situations de conservation des APL cessent avant la fin du délai maximum prévu par le code de la construction et de l'habitation. En moyenne, on constate une sortie de conservation d'environ 320 dossiers par mois, dont 300, soit en moyenne 93 %, au sens où la situation de non-décence a pris fin et le versement de l'APL a été rétabli, et seulement une vingtaine de situations dans lesquelles l'APL n'a pas été rendue une fois la période de conservation écoulée. Dans ces derniers cas, la conservation peut, dans certaines situations, être prolongée, notamment pour finir les travaux. Vous le comprenez, mesdames, messieurs les sénateurs, l'efficacité du mécanisme actuel de conservation des aides est, à notre avis, avérée. J'ajouterai que la mise en place de la conservation ne se limite pas à son caractère coercitif elle s'accompagne d'une information du propriétaire par l'organisme payeur. De façon plus globale, l'engagement de ce gouvernement est total pour lutter contre le phénomène de non-décence des logements. logements. Nous avons souhaité faire évoluer le mécanisme de conservation des aides, pour qu'il s'adapte aux politiques publiques de lutte contre le logement indécent. l'entrée en vigueur au 1 janvier 2023 et la future montée en charge du critère de non-décence énergétique, à la suite de la réforme du diagnostic de performance énergétique et aux dispositions de la loi Climat et résilience, créent une condition d'ouverture supplémentaire d'une mesure de conservation des aides. des aides. Les critères de non-décence et incidemment les causes d'ouverture d'une mesure de conservation des APL englobent la non-décence énergétique. L'obligation qui pèse sur les bailleurs a ainsi été renforcée. Pour lutter contre le fléau que constitue l'habitat indigne et dégradé, un important arsenal de procédures et de dispositifs, qui reposent la plupart du temps sur des partenariats locaux et associent notamment les collectivités territoriales, a été développé.

Pérennisés par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et reposant sur l'initiative des collectivités, ces deux dispositifs continuent de se déployer. Je tiens d'ailleurs à saluer les maires et élus locaux qui sont engagés dans cette démarche- je sais qu'ils sont nombreux. Le dispositif d'autorisation préalable de mise en de mise en location a par ailleurs fait l'objet de modifications en 2021, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à Je veux également mettre en avant le travail de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui finance l'amélioration de l'habitat des propriétaires bailleurs.

de l'année 2018, l'Anah a aussi décidé de consacrer des crédits supplémentaires, dans le cadre d'une expérimentation, à la lutte contre l'habitat indigne dans six territoires dits « d'accélération », particulièrement touchés par ces problématiques. Reconduit jusqu'en Reconduit jusqu'en 2023, ce dispositif a d'ores et déjà permis de mobiliser plus de 33 millions d'euros supplémentaires en quatre ans sur ces six départements : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l'Essonne, le Nord, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il a permis la majoration des taux de subvention pour les propriétaires occupants et bailleurs, ainsi que le financement à 100 % hors taxes des travaux d'office à la charge des communes, notamment à la suite de la prise d'arrêtés de péril. Ce dispositif, qui va se terminer dans sa forme expérimentale, fait actuellement l'objet d'une évaluation. Les résultats dégagés permettront de déterminer des axes d'action sur le champ du financement par l'Anah de la sortie d'indignité à partir de 2024. L'Anah a par ailleurs majoré depuis 2021 les crédits consacrés au financement des opérations de résorption de l'habitat indigne : ils sont passés de 15 millions d'euros à 23 millions par an. Tous les territoires engagés dans ce type d'opérations sont éligibles à ces financements. Nous aurons l'occasion, au cours du débat, d'évoquer plus particulièrement le cas des territoires ultramarins. Pour en revenir à cette proposition de loi, je le redis et vous l'avez compris, nous partageons l'objectif, mais la mesure proposée soulèverait plusieurs contraintes opérationnelles. la mutualité sociale agricole (CCMSA) -ne sont pas directement concernés par cette proposition, ils seraient néanmoins placés au coeur d'un tel dispositif, puisque la responsabilité leur reviendrait de transmettre à la Caisse des dépôts et consignations chaque ouverture de conservation des aides et, en toute logique, chaque levée de conservation. Il est d'ailleurs à noter que le système d'information de la Cnaf est actuellement surchargé, ce qui laisse envisager une difficulté réelle quant à la possibilité d'automatiser un tel signalement, sans compter la question de la sécurisation du transfert de ces données.

Enfin, à la lecture de cette proposition de loi, il est permis de s'interroger sur le potentiel effet dissuasif de la mesure proposée. En effet, la suspension du versement direct des loyers aux propriétaires pourrait inciter ces derniers à retirer leurs biens du marché de la location pour les mettre en vente. De plus, l'absence de versement du loyer résiduel peut priver certains propriétaires des ressources nécessaires pour financer la réalisation des travaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, la détermination est là, les outils sont mobilisés, et nous continuerons de lutter contre l'habitat indigne et dégradé. C'est un enjeu majeur, pour permettre à chacun, notamment aux plus modestes, de vivre dignement dans leur logement. devons faire en sorte que l'endroit où nos concitoyens se sentent à l'abri et où ils veulent se reposer après une dure journée de travail ne soit pas un logement qui les rende malades ou dans lequel ils ne supportent pas de vivre. C'est donc bien parce que le mécanisme actuel de conservation des aides est suffisant pour mettre fin aux situations de non-décence que le Gouvernement s'en remettra sur ce texte à la sagesse

En 2023, chaque Français de métropole ou d'outre-mer doit avoir accès à un logement décent et à un toit, parce que les conditions d'hébergement doivent être dignes dans un pays civilisé.

Cette situation rend encore plus insupportable l'exploitation du besoin de logement. L'habitat indigne est un fléau. Notre collègue Jean-Louis Lagourgue nous propose aujourd'hui de renforcer la lutte contre les logements non décents mis en location. En l'état actuel du droit, cela a été rappelé, les critères de décence des logements sont fixés par la loi. Il s'agit notamment de la surface et du volume minimum du logement, de l'absence de parasites et de nuisibles. Il s'agit aussi de critères destinés à la protection de la santé de l'occupant, comme une aération empêchant le développement de moisissures ou la protection du logement contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.

ou bien nous sommes d'accord pour dire qu'un logement mis en location doit satisfaire aux critères de décence fixés par la loi, auquel cas les mesures portées par la proposition de notre collègue ne constituent que la poursuite de la logique qui sous-tend le droit actuel ; ou bien nous considérons qu'un logement non décent peut valablement continuer à être une source de profits pour des bailleurs peu scrupuleux. « Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre », selon le cardinal de Richelieu. Nous pensons donc qu'un logement non décent, c'est-à-dire une mise en location illégale, ne doit pas générer de profit.

ils ne sont pas tous petits, loin de là -, mais suffirait-il d'être un petit bailleur pour être exonéré du respect de la loi ? Par ailleurs, en tout état de cause, le propriétaire bailleur conserve toujours la capacité de vendre son bien s'il ne peut en assumer la décence.

cette proposition est néanmoins le signe que l'île rencontre en matière de logement un problème majeur, qui appelle une réponse rapide. Jean-Louis Lagourgue a déposé un amendement pour que cette proposition de loi ne s'applique qu'à titre expérimental et temporaire sur le territoire de La Réunion. L'expérimentation permettrait à la fois d'agir rapidement et de recueillir des données utiles au perfectionnement du dispositif. À l'inverse, ne rien faire reviendrait à prendre encore du retard dans un domaine où l'urgence est déjà là. La loi fixe déjà les critères de la décence des logements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout comme l'habitat insalubre et l'habitat indigne, le chantier de l'habitat non décent est gigantesque. Comme le soulignait notre rapporteur, sur l'ensemble du territoire français, au moins 420 000 logements seraient indignes, dont 110 000 dans les départements et régions d'outre-mer, particulièrement confrontés à ces difficultés. Contrairement aux procédures relatives à l'indignité, à l'insalubrité ou au péril, qui relèvent des autorités administratives, la lutte contre la non-décence relève exclusivement d'une action privée, celle du locataire contre le bailleur.

Je ne reviendrai pas en détail sur le dispositif actuel, car vous l'avez toutes et tous à l'esprit. L'article unique de cette proposition de loi tend à consigner le reste à charge du loyer auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le locataire continuerait de payer le loyer, mais celui-ci ne serait plus versé au bailleur. Cette mesure semble, de prime abord, aller dans le bon sens pour répondre à l'objectif indispensable de lutte contre la non-décence des logements. L'examen en commission a toutefois mis en avant un certain nombre d'écueils et le manque d'opérationnalité du dispositif. également estimé que le dispositif actuel de consignation du montant des APL fonctionnait dans la majorité des cas pour que les travaux soient engagés. Plus de 95 % des procédures aboutiraient à une remise en état dans les dix-huit mois impartis, selon les services de l'État.

En effet, nombre de propriétaires rencontrent eux-mêmes des difficultés financières et peinent à financer les travaux, comme le démontrent régulièrement les rapports de la Fondation Abbé Pierre. Encore une fois, l'accompagnement des bailleurs est l'un des sujets essentiels Le risque que ce nouveau mécanisme rende l'actuel plus complexe et moins lisible a aussi été souligné. Pour l'instant, après le signalement à la CAF, le locataire n'a aucune démarche supplémentaire à effectuer, puisque la CAF procède d'elle-même à la retenue des allocations de logement. Le dispositif proposé est plus complexe. Il introduit une procédure active de consignation du reste à charge. Une mauvaise compréhension du dispositif pourrait conduire une partie des locataires vers des situations d'impayés de loyer, qui pourraient déboucher sur leur expulsion. Par ailleurs, le texte n'aborde pas la question épineuse du sort des reliquats des loyers qui resteraient consignés une fois la période de blocage des aides révolue. Qu'adviendrait-il de ces sommes ?

le locataire aura donc tout intérêt à avoir saisi un juge pour obliger son bailleur à réaliser les travaux nécessaires ou à faire réduire son loyer. Cela soulève la question de l'opportunité de saisir le juge. Le plus efficace serait donc de prévoir une procédure simplifiée pour obtenir plus rapidement une décision de justice. Se pose également la question de la possibilité de remise en location du logement si les travaux ne sont toujours pas effectués, mais le texte n'y répond pas non plus. Compte tenu de ces éléments, la question de l'opérationnalité du dispositif est posée et sa plus-value n'est pas évidente, dans la mesure où il ne tend pas à améliorer le sort du locataire de manière significative. Il est peut-être même contre-productif, car le risque que le dispositif fragilise les propriétaires modestes et les locataires semble réel, à La Réunion comme en métropole.

production massive de logements sociaux, à l'encadrement des loyers en secteurs tendus, à l'augmentation des APL, à la garantie universelle des loyers, à l'intensification de la prévention des expulsions locatives, renforcement des moyens pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et, bien sûr, à un réel accompagnement humain et financier des propriétaires pour la rénovation de leur logement. Il convient également de communiquer plus efficacement auprès des publics concernés sur les différents dispositifs existants qui s'offrent à eux pour la réhabilitation de leur logement.

la proposition de loi que notre assemblée examine ce matin vise à augmenter la contrainte qui pèse sur les bailleurs, afin de les inciter à procéder aux travaux de mise en décence et de rénovation des logements loués à des allocataires d'aides personnelles au logement. Si le sujet des logements non décents et insalubres ou indignes n'est pas nouveau, force est de constater que celui-ci persiste en métropole comme dans les outre-mer. Aujourd'hui, le constat est sans appel : il y aurait 420 000 logements indignes au sein du territoire national, dont 110 000 dans les outre-mer, selon les chiffres cités par un récent rapport de la délégation sénatoriale La Réunion est particulièrement affectée par ces dégradations de logement, ce qui explique, sans aucun doute, le dépôt de cette proposition de loi par notre collègue, M. Jean-Louis Lagourgue, sénateur de La Réunion, reprend ainsi le texte déposé voilà un an, en février 2022, par l'ancien député de ce même territoire, M. David Lorion. Introduite par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU, la notion de non-décence ne concerne, en droit, que le logement locatif. L'objectif du législateur était clairement de préciser l'obligation faite aux bailleurs de délivrer un logement en bon état et qui réponde à des normes minimales en matière de confort. Par conséquent, pour être qualifié de décent, un logement doit notamment présenter une surface minimale, une absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, une absence d'animaux nuisibles et de parasites, ainsi que la mise à disposition de certains équipements nécessaires à le rendre habitable- rendre habitable- le chauffage, l'électricité ou le système d'évacuation des eaux usées. Toutefois, depuis le 1 janvier 2023, en application de la loi Énergie et climat, les logements locatifs doivent également répondre à des critères de performance énergétique pour pouvoir être qualifiés de « décents ». Ces critères seront progressivement durcis jusqu'en 2034, date à laquelle l'ensemble des logements classés E, F ou G ne pourront plus être loués. Les transitions écologiques et énergétiques nous imposent de légiférer. Nous avons commencé le travail et nous le poursuivrons ! Autrement dit, mes chers collègues, notre groupe partage bien évidemment l'objet affiché par ce texte, qui vise à protéger davantage les locataires face au fléau que représentent les logements non décents. Cela étant, je constate à mon tour que le dispositif proposé dans le texte est inadapté et qu'il risque de complexifier et d'aggraver la situation des locataires. locataires. Le mécanisme proposé dans l'article unique est inadapté et inopérant. Il est inadapté, car faire en sorte que le loyer soit désormais non plus versé au bailleur, mais consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations soulève des interrogations sur le plan opérationnel, en particulier pour les organismes payeurs que sont la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA). Si ces organismes ne sont pas directement concernés, ils seraient néanmoins placés au coeur coeur du mécanisme, puisqu'il leur reviendrait de transmettre à la Caisse des dépôts et consignations chaque ouverture de conservation des aides et, en toute logique, chaque levée de la conservation. Compte tenu de la surcharge d'activités actuelle du système d'information de la Cnaf, nous pouvons craindre une réelle difficulté quant à la possibilité d'automatiser un tel signalement, sans compter la question de la sécurisation du transfert de ces données et celle du coût que cela représenterait. Le dispositif est donc inadapté, mais il est également inopérant, car on peut s'interroger sur le potentiel effet dissuasif de la mesure proposée. Je rappelle que la procédure actuelle de retenue des allocations de logement démontre une certaine efficacité, puisque, selon les services de l'État, plus de 95 % des dossiers aboutissent à une remise en état dans les délais impartis. Contrairement à la situation en métropole, la procédure existante concerne également les bailleurs sociaux dans les outre-mer. Or ces derniers semblent affirmer que la privation du reste à charge du loyer n'influerait en rien sur leur diligence à traiter les cas de non-décence. De plus, l'absence de versement du loyer résiduel pourrait priver des propriétaires, au moins les plus modestes, des ressources nécessaires pour financer la réalisation de travaux. Ce sont autant de raisons qui démontrent que le dispositif du texte est inadapté et inopérant. ailleurs, le mécanisme risque d'entraîner des conséquences non négligeables sur les locataires. Pour l'instant, après un signalement à la Cnaf, les locataires n'ont aucune démarche à effectuer pour que les allocations de logement cessent d'être versées aux bailleurs. Introduire une procédure active de consignation du reste à charge pourrait amener une partie des locataires à cesser de payer leur loyer, ce qui les exposerait à une expulsion, tout à fait légale, à la demande du propriétaire. Pis encore, la suspension du versement direct des loyers aux propriétaires pourrait inciter ces derniers à retirer leurs biens du marché de la location pour les mettre en vente. Mes chers collègues, si l'intention de l'auteur de ce texte est louable, le dispositif me semble inadapté à l'objectif qui fait sans doute consensus au sein de cette assemblée, à savoir un meilleur accompagnement des bailleurs, dans l'intérêt des locataires et de nouvelles solutions face à la dégradation des logements, qui dépasse largement le seul champ du logement non décent. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI s'abstiendra sur ce texte. La parole

600 000, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui ne saurait être accusée d'excès, compte tenu des situations dramatiques qu'elle étudie et suit de près. Selon ce même rapport, rien ne permet d'indiquer une quelconque évolution positive en 2022, et aucune dynamique n'a été lancée pour les années à venir. Dans les territoires d'outre-mer, la situation est particulièrement critique. Selon le rapport d'information sénatorial sur la politique du logement en outre-mer, près de 13 % du parc sont jugés indignes.

Un chiffre semble fiable : 600 000 enfants vivraient dans ces conditions aujourd'hui dans notre pays. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à mieux protéger les locataires bénéficiant d'une allocation logement et vivant dans des habitats considérés comme non décents.

Ce délai doit permettre au bailleur d'effectuer les travaux nécessaires pour rendre le logement apte à la location. Si nous adoptions cette proposition de loi, le locataire d'un logement indécent verserait le loyer résiduel non plus au bailleur, mais à la Caisse des dépôts et consignations. De ce fait, le bailleur ne percevrait plus aucune somme tant que le logement ne répondrait pas aux normes de décence. Si nous comprenons bien l'intention qui se trouve derrière cette proposition, nous ne pouvons manquer de formuler plusieurs réserves. En premier lieu, il existe déjà des procédures permettant d'inciter le bailleur à effectuer des travaux de réhabilitation d'un logement non décent. Comme l'a rappelé en commission Mme le rapporteur, contrairement aux procédures relatives à l'indignité, à l'insalubrité ou au péril, qui relèvent des autorités administratives, la lutte contre la non-décence relève exclusivement d'une action privée, celle du locataire contre le bailleur. Si ce dernier refuse d'exécuter les travaux de remise en état d'un logement en situation de non-décence, le locataire peut en effet saisir le juge. Le juge peut notamment ordonner l'exécution des travaux, assortie d'une éventuelle réduction du montant du loyer pour toute la durée pendant laquelle le logement demeure non décent. Cette procédure a concerné 2 647 situations en 2017 et 4 079 en 2019. Le chiffre est en augmentation, ce qui signifie bien que les locataires, mieux informés sur leurs droits, n'ont pas hésité à les faire valoir auprès des autorités compétentes. La grande majorité des travaux ont été effectués dans les dix-huit mois par les propriétaires. lieu, le dispositif proposé par nos collègues du groupe Les Indépendants - République et Territoires pourrait entraîner des conséquences négatives, sans répondre pour autant de manière efficace à la lutte contre les logements dégradés.

Depuis la loi Climat et résilience, les logements doivent présenter une performance énergétique minimum. Cela se traduit par l'interdiction de louer les logements les plus énergivores à compter du 1 janvier 2023 et par l'interdiction progressive de louer les logements de catégorie G

Or force est de constater que la politique menée ces dernières années ne produit pas les effets escomptés, car les aides sont mal ciblées. Rémi Cardon sont mal ciblées. Rémi Cardon et moi avons déposé une proposition de loi pour recentrer l'effort budgétaire du pays sur l'éradication des passoires thermiques et engager une stratégie de rénovation plus

Les raisons sont simples. Trop peu de personnes s'engagent dans un parcours de rénovation. Près de la moitié des ménages résidant en passoire thermique ont des revenus modestes, voire très modestes. Quelque 37 % de ces logements sont occupés par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Toujours selon la Fondation Abbé Pierre, le reste à charge des plus modestes serait actuellement de l'ordre de 39 % pour une rénovation globale, ce qui est bien trop important pour les familles les plus précaires, y compris dans le cadre du prêt avance rénovation mis en place par le Gouvernement,

urgence, également, car les logements les plus énergivores vont disparaître du marché de la location, faute de rénovation. Cette interdiction est entrée en vigueur au 1 janvier 2023 pour les logements de classe G, c'est-à-dire pour ceux qui ont une consommation supérieure à 450 Il y a urgence, enfin, à prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins, à promouvoir les techniques les mieux adaptées et à faciliter le recours à des matériaux de construction et de rénovation produits et utilisés localement. Ainsi, plutôt que de confisquer, pour ainsi dire, les revenus locatifs des propriétaires, nous pensons qu'il est préférable de mieux les accompagner. Il est nécessaire que les citoyens perçoivent enfin les signes concrets et positifs de la transition énergétique. Celle-ci est encore trop souvent perçue comme inefficace et inégalitaire. Notre politique climatique et énergétique doit comporter une stratégie de rénovation des logements et de lutte contre la précarité énergétique plus performante et plus inclusive. Notre priorité devrait être de sortir les 5,6 millions de ménages de la précarité, qu'ils soient propriétaires ou

La proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui est audacieuse. Elle a le mérite de poser clairement le problème du mal-logement et d'y apporter des éléments de réponse. En vous attaquant aux logements non décents, vous soulevez aussi, et peut-être même surtout, la question des passoires thermiques. Plusieurs catégories de logements seront progressivement interdites à la location ; tant mieux pour les locataires et pour la lutte contre le gaspillage d'énergie ! Cela concerne d'abord les logements G+, dès cette année, puis G, à partir de 2025, F en 2028, et ainsi de suite. Nous sommes tout à fait convaincus qu'il faut développer des mesures fortes contre ces passoires thermiques. Les situations sont très inégales sur le territoire, mais elles sont trop nombreuses. Il sera nécessaire d'agir en profondeur pour mieux isoler les logements et mieux protéger les locataires. 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique. Cet enjeu doit être prioritaire. Tous les outils pour mesurer les performances énergétiques des logements ne sont pas toujours concordants. Il est nécessaire d'affiner quelque peu pour qu'aucun logement ne sorte des radars ou ne soit intégré à la mauvaise catégorie. Il y a un besoin réel et urgent de vérifier la fiabilité de la classification et de déterminer des outils et un référentiel qui soient identiques, quelles que soient la localisation du logement

du multipropriétaire qui empoche de nombreux loyers sans jamais mettre un euro dans l'entretien ou l'isolation du logement. Il faut aussi faire la part des choses avec les bailleurs sociaux, dont les finances ont été durement ponctionnées, notamment avec la réduction de loyer de solidarité Pour les propriétaires de bonne foi, comme pour les bailleurs sociaux, la réponse selon laquelle il faudrait bloquer leurs ressources pour qu'ils fassent les travaux est un peu contradictoire. C'est à peu près le même niveau de réflexion que de dire que l'on bloque les APL pour les locataires qui n'arrivent plus à payer leur loyer

Ce sera bon pour les finances de nos concitoyens comme pour notre planète. Il faudra donc, avant tout, proposer des moyens aux bailleurs, publics comme privés, pour que chacun vive dignement dans un logement décent. Telle est notre préoccupation première

lui, vise à donner au juge la responsabilité de suspendre le bail et de décider du montant de loyer versé, le temps que le propriétaire fasse les travaux de mise aux normes, avec une prise différée du bail pour empêcher la mise à la rue du locataire qui aurait fait valoir ses droits. Nous nous exprimerons aussi au sujet des logements décents, plus particulièrement des passoires thermiques, dans le cadre de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Pour l'heure, votre proposition de loi demeure incomplète, peut-être même contre-productive, et surtout cantonnée à une partie du territoire français, ce qui est à notre avis regrettable. C'est pourquoi, en l'état, notre groupe s'abstiendra. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure où la vie n'a jamais été aussi chère et où la précarité ne cesse d'augmenter, le logement demeure la première dépense contrainte de nos concitoyens, à hauteur de 30 % à 40 % de leur budget. Nous devons plus que jamais nous saisir du sujet et le mettre à l'ordre du jour pour agir concrètement afin d'améliorer le quotidien des Français. Toutes les initiatives allant dans ce sens sont à saluer. Je tiens donc à remercier notre collègue Jean-Louis Lagourgue et les autres signataires de cette proposition de loi, qui ont ainsi permis de relancer le débat sur la situation du logement dans notre pays, un sujet qui préoccupe tant de nos concitoyens. Je salue également les apports précieux de la rapporteure Micheline Jacques et de la commission des affaires économiques ; ils rappellent tout l'intérêt et toute la vitalité du travail parlementaire. Toutefois, avec mes collègues de l'Union Centriste, nous considérons que ce texte n'est pas abouti, à ce jour, et partageons la position de la rapporteure. Nous souscrivons évidemment à la volonté de protéger plus efficacement les locataires confrontés à des bailleurs malveillants, mais nous tenons également à ce que les propriétaires les plus modestes, qui sont, de surcroît, le plus souvent de bonne foi, ne soient pas pénalisés par un dispositif qui risquerait, en l'état, d'être trop rigide. Priver un petit bailleur du loyer qu'il perçoit pourrait en effet lui faire perdre une part importante de ses revenus, qui n'excèdent parfois pas ceux de ses locataires. Cela pourrait aussi, tout simplement, l'empêcher de procéder aux travaux nécessaires à la rénovation du logement, ce qui irait à l'encontre de l'objectif des auteurs de la proposition de loi. De plus, la procédure de constat en non-décence, bien que trop peu usitée, a fait preuve de son efficacité et nous manquons de données pour évaluer d'éventuels dysfonctionnements. Enfin, le déficit que connaît notre pays en matière d'offre de logements nous astreint à faire preuve de pragmatisme et de nuance. Certains propriétaires ne seront jamais prêts à louer s'ils craignent que la mise en location de leur bien représente,, une charge plutôt qu'une source de revenus. Or nous avons plus que jamais besoin de nouveaux bailleurs. C'est en ayant ces éléments à l'esprit que, avec une grande majorité du groupe Union Centriste, nous suivrons la rapporteure et la commission en votant contre l'adoption de ce texte. Je veux profiter du reste du temps qui m'est imparti pour mettre l'accent sur les urgentes priorités qui doivent être les nôtres en matière de logement. Les chiffres du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre nous rappellent la réalité brutale du mal-logement dans notre pays. Aujourd'hui en France, on compte 330 000 sans-abri et 4,1 millions de personnes mal logées ; plus de 12 millions de personnes se trouvent en situation de fragilité en matière de logement. Or les personnes qui paient le plus lourd tribut au mal-logement, ce sont, comme souvent, les femmes. Il est plus difficile pour une femme, et plus encore pour une mère célibataire, de sortir du mal-logement renforce la précarité des femmes et les expose, plus que les hommes, au risque de violences sexuelles. Le logement reste malheureusement le creuset des inégalités dans notre pays. Face à cette situation, il serait faux de dire que le Gouvernement est demeuré passif : 440 000 personnes sont sorties de l'hébergement d'urgence ou du sans-abrisme grâce au plan Logement d'abord au cours du dernier quinquennat 250 000 logements sociaux ont été construits entre 2021 et 2022 ; enfin, 6,7 milliards d'euros ont été consacrés par le plan France Relance à la rénovation des logements privés et sociaux, des bâtiments publics et des locaux des PME-TPE. pour atteindre les objectifs ambitieux auxquels nous astreint la situation du logement dans notre pays, ces efforts doivent être poursuivis et complétés. L'offre de logements demeure en effet très insuffisante au regard des besoins croissants de la population, en particulier dans les territoires qui connaissent les tensions les plus fortes. Cela s'explique, tout d'abord, par la raréfaction du foncier. Nous manquons de terrains constructibles et nous devrons veiller à ce que l'objectif de « zéro artificialisation nette » des sols en 2050, le fameux ZAN, ne fasse pas peser de contraintes trop lourdes sur la construction de logements neufs. Je salue à ce titre l'excellent travail réalisé par la commission spéciale présidée par Valérie Létard autour de la proposition de loi dont nous débattons cette semaine. Ce sont des signes forts envoyés aux acteurs de nos territoires. En outre, la construction et l'amélioration des logements sont compliquées par le foisonnement des normes qui les encadrent. Entre 2002 et 2022, le code de l'urbanisme est passé de 1 584 à 3 542 pages. La prolifération des normes augmente le coût de la construction et peut en limiter le volume ; parfois, ces normes sont tout simplement absurdes. Je me réjouis à ce propos que la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, présidée par notre collègue Françoise Gatel, organise ce matin même les États généraux de la simplification. La crise de l'offre est enfin celle de la location. Il importe à ce titre que les bailleurs soient accompagnés dans la rénovation de leurs logements, afin que les obligations de performance énergétique auxquels ils sont soumis ne représentent pas une charge trop lourde et désincitative.

C'est l'une des missions du Parlement que d'évaluer et de contrôler les politiques publiques. Mes chers collègues, gardons toujours à l'esprit ces mots de l'abbé Pierre : « Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. » Le logement est un sujet complexe, qui fait intervenir de très nombreux acteurs et soulève des problématiques variées, qu'elles soient de nature économique, sociale, ou environnementale. Je souhaite que l'initiative de Jean-Louis Lagourgue, à défaut de constituer à ce stade une réponse viable à la problématique du mal-logement, marque le début d'un vrai débat de fond sur ces questions chères aux Français. La parole

C'est ainsi qu'on garantit que chacun pourra satisfaire l'un des besoins les plus essentiels et qu'on lui apporte sécurité physique et préservation de la santé. La lutte contre le mal-logement doit donc constituer une priorité nationale, quel que soit le territoire concerné.

À La Réunion, territoire cité dans l'exposé des motifs de ce texte, 18 000 logements seraient concernés ; la tendance est à la hausse. Les chiffres concernant la non-décence sont plus complexes à obtenir. La présente proposition de loi procède à une légère modification de la loi en vigueur, de manière à inciter le propriétaire d'un logement non décent pour lequel des allocations de logement sont versées à réaliser les travaux de mise en conformité au plus vite. Elle dispose que le locataire consigne le montant du loyer qui lui incombe- déduction faite des allocations -auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), plutôt que de le verser au bailleur. Il apparaît que la mise en place de la suspension du versement des allocations de logement au propriétaire pendant ce délai, limité à dix-huit mois, mais prolongeable de six mois, a porté ses fruits. Le droit en vigueur serait donc suffisamment dissuasif pour provoquer la remise en état du bien. En effet, le taux de libération des allocations serait de 95 %, soit une très forte effectivité. a par ailleurs exprimé ses craintes quant au caractère contre-productif du dispositif proposé, qui retirerait aux propriétaires modestes les moyens financiers nécessaires à la réalisation des travaux. Or, rappelons-le, ces derniers peuvent donner lieu à des aides à la rénovation. Encore faut-il que le locataire signale à la caisse d'allocations familiales l'état de non-décence de son logement. C'est tout le problème lorsque la demande est loin de satisfaire l'offre. Le locataire est prêt à tout accepter pour dormir sous un toit. Que le dispositif ne soit pas adapté, soit ! Mais l'argument selon lequel il enverrait au locataire le signal de ne pas payer le loyer ne nous a pas convaincus. Si l'on exclut une minorité de mauvais payeurs, la principale préoccupation des locataires et notamment des plus modestes d'entre eux est de parvenir à régler le loyer, par peur de l'expulsion. D'ailleurs, il aurait été intéressant de disposer de chiffres plus précis quant aux délais de réalisation des travaux. Est-ce qu'ils sont majoritairement réalisés dans un délai de 6, 12, 18 ou 24 mois ?

Bien que les deux tiers des logements non décents soient traités au bout d'un an dans le cadre de cette procédure, son expérimentation à La Réunion, proposée au travers de l'amendement déposé par M. Lagourgue, pourrait nous éclairer sur ce point.

L'excellent rapport sur ce sujet de la délégation sénatoriale aux outre-mer, dont notre collègue Micheline Jacques était l'un des auteurs, pointe un certain nombre de défaillances. Si le contrôle de la qualité des nouvelles constructions demeure déficient, on alimente la machine à produire de l'habitat indigne. Il est ahurissant de constater que la moitié des habitants de La Réunion affrontent des problèmes d'humidité dans leur domicile. La multiplication des malfaçons, notamment sur des constructions de moins de dix ans, alors même que les règles se renforcent, doit être rapidement réglée par les pouvoirs publics. Nous faisons donc face à un défi à la fois quantitatif et qualitatif. Où en est-on des plans logement outre-mer ? Après l'échec du premier, le bilan en attente du deuxième et l'abandon du troisième, quelles solutions sont envisagées ? J'espère, monsieur le ministre, que, après le débat qui s'est tenu en janvier dernier au sein de cet hémicycle, vous pourrez nous donner plus de précisions sur les réponses qui seront apportées à la crise du logement en outre-mer, en particulier à La Réunion, mais aussi, en général, sur l'ensemble du territoire.

je remercie notre collègue Jean-Louis Lagourgue et le groupe Les Indépendants de donner, ce matin, l'occasion à notre assemblée de faire un point sur la lutte contre le logement indécent dans notre pays et, plus particulièrement, outre-mer. C'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur et sur lequel je me suis beaucoup investie, avec la commission des affaires économiques et sa présidente Sophie Primas, notamment après le drame de la rue d'Aubagne, survenu le 5 novembre 2018, très présent encore dans nos mémoires. Le logement est un bien de première nécessité, avons-nous coutume de répéter. C'est aussi un droit et un élément central de notre pacte républicain. C'est l'abri de la famille, la protection de la vie privée, une possibilité d'épanouissement personnel et, normalement, une garantie d'égalité, car grandir dans un logement délabré diminue les chances de réussite et même l'espérance de vie. Mais ce droit est également un combat. Il nous mobilise, quel que soit notre groupe politique. Ce combat se fonde sur des principes simples- l'égalité, la justice et l'humanité -, mais il se décline dans des réalités compliquées. Malheureusement, il n'y a pas de martingale, pas de cause ou de responsable uniques, pas de baguette magique pour une solution immédiate. Cette tension, nous la ressentons aujourd'hui en examinant la proposition de loi qui nous est soumise. La rapporteure de la commission, Micheline Jacques, dont je tiens à saluer le travail de fond, a osé affronter la complexité de la lutte contre l'habitat indécent et ne s'est pas contentée de solutions séduisantes, mais mal adaptées.

S'appuyant sur le rapport d'information de juillet 2021 de notre délégation aux outre-mer, dont Micheline Jacques était déjà l'un des auteurs, Jean-Louis Lagourgue souligne qu'environ 13 % des logements seraient considérés comme indignes dans les départements et régions ultramarins, soit 110 000 sur 900 000. C'est certainement un problème central et urgent. Pour y porter remède, l'auteur de la proposition de loi

À première vue, on peut être séduit par la solution qui désigne un coupable et un seul : le bailleur ! C'est malheureusement trop simple. Le rapport de la commission a démonté cette fausse évidence. On doit relever tout d'abord que le droit actuel, qui prévoit la retenue des APL lorsque le locataire fait valoir une situation d'indécence, est efficace dans 95 % des cas. Il permet donc, d'ores et déjà, d'apporter les solutions attendues. Aller plus loin en retirant toute ressource aux propriétaires bailleurs aurait donc une dimension plus punitive qu'incitative, approche qui n'est pas justifiée par les faits. À La Réunion, la Fondation Abbé Pierre a estimé que la majorité des logements problématiques appartenaient à des propriétaires modestes dont les conditions de vie sont similaires à celles de leurs locataires. le sait, à l'échelle nationale, un tiers des propriétaires ne sont pas imposables et deux tiers n'ont qu'un seul bien à louer, souvent pour compléter une retraite. Par ailleurs, à La Réunion, de nombreux logements indécents sont des logements sociaux ; leur caractère indécent est notamment dû à des problèmes d'infiltrations. On se rend alors compte qu'il s'agit moins d'un conflit de classes entre propriétaires et locataires que d'un problème plus structurel de qualité du bâti, y compris pour les constructions récentes. Utiliser l'outil de l'indécence des logements, c'est aussi faire reposer le poids de la résorption de l'habitat indigne sur les seuls locataires, dont on sait que beaucoup hésiteront à lancer une procédure face au risque de ne pas disposer d'un autre logement et de perdre le bénéfice des APL après les dix-huit mois de suspension s'ils demeurent dans le logement. Par ailleurs, centrer la lutte contre l'habitat indigne sur les seuls locataires, c'est laisser de côté un pan important du sujet : les nombreux propriétaires

En outre-mer, l'habitat informel, ou spontané, est un sujet souvent important, mais il ne résulte pas de difficultés dans les relations entre propriétaires et locataires. Enfin, les problèmes de logement indigne outre-mer, et plus particulièrement à La Réunion, ont un caractère structurel qui dépasse largement les défaillances d'entretien des logements. Le rapport de la commission, sur la base des témoignages des services de l'État, mais aussi des associations de locataires et des bailleurs sociaux, pointe des malfaçons récurrentes, une formation et une qualification insuffisantes des professionnels et des matériaux inappropriés. Ainsi, beaucoup d'immeubles récents, encore sous garantie décennale, seraient aujourd'hui problématiques. Certains de ces défauts pourraient s'expliquer par un usage mal contrôlé des possibilités d'investissement défiscalisé. Aussi, plutôt que de mettre en cause les seuls propriétaires bailleurs, le problème de l'habitat indigne outre-mer ne pourra trouver de solutions qu'à la suite d'une analyse multifactorielle de ses différentes causes, d'autant que ces départements font face à des risques sismiques et climatologiques spécifiques. je regrette que l'auteur de la proposition de loi n'ait pas accepté la proposition d'un renvoi en commission, qui aurait permis de procéder à cette analyse conjointement avec la délégation aux outre-mer. C'est pourtant la solution que nous avions trouvée sur la proposition de loi déposée par notre collègue Bruno Gilles à la suite du drame de la rue d'Aubagne. Nous avions pu mener un travail en profondeur et faire adopter la proposition de loi modifiée quelques mois plus tard. Une expérimentation du dispositif évoqué dans la seule île de La Réunion

par son auteur. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l'article unique de la proposition de loi initiale.

Madame le rapporteur, chère collègue ultramarine, je pense que vous comprenez notre situation. Je veux croire que vous ne vous opposerez pas à la demande de la quasi-totalité des parlementaires de La Réunion, pour leur territoire et leurs concitoyens. Quel est l'avis de la commission ? Le présent amendement

une période courant jusqu'au 31 décembre 2026, à titre expérimental. Toutefois, les motifs qui font douter de l'adéquation du dispositif proposé à l'objectif de ses auteurs sont tout aussi valables à La Réunion que sur le reste du territoire national.

durcir ? Concernant le risque de fragilisation des propriétaires modestes, je me reporte à un récent rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui soulignait justement le manque de ressources des bailleurs privés de La Réunion pour réhabiliter leurs logements. J'ajoute que, si les critères de performance énergétique ne s'appliquent pas pour l'instant dans les outre-mer, ils y entreront progressivement

de la Deal de La Réunion. Je comprends la tentation de l'expérimentation, face aux situations ubuesques dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais, je le répète, le dispositif n'est pas efficient et les risques d'effets de bord sont réels, à La Réunion comme ailleurs. En outre,